visant à faire face à la situation économique sans précédent à laquelle la France est confrontée, comme tous les autres sur la planète. La situation économique dans laquelle nous nous trouvons- j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises -n'a pas d'autre équivalent que la grande récession de 1929 par la violence du choc que nous avons connu. Nous maintenons donc notre prévision de récession de moins 11 % du PIB pour 2020. Nous disposons aujourd'hui de premiers indicateurs positifs, qui montrent que les mesures que nous avons prises avec le Président de la République et le Premier ministre ont permis de restaurer une confiance et d'engager un certain nombre de décisions économiques positives. Je pense à la consommation des ménages, qui se maintient. Je pense aussi aux créations d'entreprise, qui ont retrouvé en juin 2020 leur niveau de juin 2019. Tous ces indicateurs positifs ne modifient pas pour le moment notre prévision de croissance pour 2020, mais ils nous encouragent à poursuivre et à intensifier nos efforts de soutien à l'économie. Je veux profiter de cette prise de parole pour redire à tous nos compatriotes que, depuis le premier jour, avec le Président de la République et le Premier ministre, nous avons répondu présents pour soutenir les entreprises et pour protéger les salariés. Aussi longtemps que durera cette crise économique, nous serons présents pour soutenir les entreprises et pour protéger les salariés. Je veux également profiter de cette intervention pour rappeler les différentes mesures que vous avez adoptées et qui nous ont permis d'amortir le choc économique qui est tombé sur la France.

300 milliards d'euros ont été engagés au travers des prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, un demi-million d'entreprises ont bénéficié de ces prêts garantis pour un montant de 100 milliards d'euros,

30 milliards d'euros ont financé l'activité partielle de millions de salariés. Nous avons fait un choix politique majeur : défendre l'emploi au prix d'un endettement accru de la France, parce que nous estimons qu'il coûte moins cher de protéger l'emploi au prix d'un endettement que d'aboutir à des drames sociaux partout sur le territoire français. Le fonds de solidarité que nous avons prévu pour les petites entreprises et pour les indépendants a bénéficié à 1,7 million de très petites entreprises, qui ont reçu plus de 5 milliards d'euros.

avec un deuxième projet de loi de finances rectificative. Elle continue aujourd'hui avec ce troisième projet de loi de finances rectificative, qui, comme les deux premiers, vise l'objectif d'adapter nos réponses à la réalité de la situation économique. Elle se poursuivra enfin, dès la fin de l'été, grâce à un plan de relance de 100 milliards d'euros, qui sera présenté par le Président de la République et le Premier ministre.

Il n'y aura donc pas de quatrième projet de loi de finances rectificative, ni de loi ordinaire supplémentaire. Nous avons privilégié la simplicité, la la cohérence et la rapidité en inscrivant toutes ces nouvelles mesures dans le projet de loi de finances pour 2021, avec un seul objectif : répondre le plus vite possible aux entreprises, aux filières industrielles et aux salariés qui s'inquiètent pour leur emploi.

S'agissant du texte que nous examinons aujourd'hui, pour simplifier la présentation, je dirai qu'il repose sur deux volets essentiels. Le premier volet, c'est le soutien aux entreprises. Nous avons fait le choix de cibler notre soutien sur les entreprises et les secteurs les plus fragilisés par la crise, grâce à une série de plans sectoriels. Dans l'aéronautique, l'activité partielle de longue durée, par exemple, permettra à des entreprises comme Safran d'éviter tout licenciement dans les mois à venir. Je salue d'ailleurs l'accord qui a été conclu chez Safran ; il montre que, lorsque chefs d'entreprise et salariés peuvent s'entendre avec les représentants syndicaux, on sauve l'emploi sans amoindrir la compétitivité de l'entreprise. Le texte de loi propose aussi un certain nombre de mesures pour le petit commerce, qui a été particulièrement touché par cette crise ; vous le constatez tous sur le territoire et dans les communes dont vous êtes les êtes les élus. Quelque 100 foncières seront déployées partout en France à l'aide de la Banque des territoires, pour rénover 6 000 petits commerces. La Banque des territoires achètera donc des locaux, elle les réunira lorsque ce sera nécessaire, engagera des frais de rénovation thermique puis les louera à des commerçants un tarif préférentiel de façon à revitaliser le commerce qui a été très durement touché, en particulier dans les communes rurales, par la crise économique. Pour les entreprises technologiques, 500 millions d'euros ont été réservés, pour éviter que des start-up à fort potentiel ne fassent faillite uniquement à cause d'un manque

du plan pour l'industrie automobile présenté par le Président de la République nous ont permis de relancer une industrie qui était en situation extraordinairement fragile à cause de la crise économique. Les bonus pour l'achat d'un véhicule propre et la prime à la conversion ont connu un immense succès. Nous sommes un des seuls pays européens dont le nombre d'immatriculations a augmenté en juin 2020 par rapport à juin 2019.

et les véhicules hybrides rechargeables, afin d'atteindre notre objectif stratégique de décarbonation du parc automobile français. Par ailleurs, au-delà de ces plans de relance sectoriels, et toujours au titre de ce premier volet de soutien aux entreprises, nous voulons continuer à soutenir la trésorerie des entreprises, des entreprises, car elle est aujourd'hui la plus menacée et la plus en difficulté. Deux chantiers que nous avons lancés il y a maintenant plusieurs semaines vont être prolongés et renforcés. Le premier est celui des reports de charges. Vous le savez, nous avons déjà fait beaucoup pour reporter un maximum de charges sociales et fiscales : 35 milliards d'euros au total depuis mars dernier, dont 22 milliards d'euros de reports de charges sociales et 13 milliards d'euros de reports de charges fiscales. À ces reports, nous avons ajouté des mesures inédites d'exonération de cotisations sociales pour les secteurs les plus touchés par la crise : pour l'hôtellerie, pour la restauration, pour la culture, pour l'événementiel, pour le tourisme, pour le transport aérien et pour les secteurs qui sont dépendants du transport aérien, nous avons annulé près de 4 milliards d'euros de cotisations sociales.

ils l'ont obtenu pour préserver l'activité et l'emploi. Nous voulons compléter ce dispositif, car nous avons parfaitement conscience qu'il faut continuer à tirer le fil de l'étalement ou des reports de charges sociales et fiscales, pour éviter qu'un mur

mois et que ce dispositif soit accessible à toutes les PME et toutes les TPE, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit la baisse de chiffre d'affaires qu'elles ont connue. plus, nous proposons que l'entreprise n'ait pas à solliciter cet étalement : elle n'aura qu'à présenter une demande au service des impôts qui, au vu de son ratio d'endettement, lui indiquera la durée possible d'étalement des charges de manière automatique.

à l'inquiétude des entreprises et nous allégeons leur trésorerie. Une deuxième inquiétude m'est relayée depuis plusieurs semaines- vous savez que j'ai toujours eu à coeur d'entendre ce qui se disait auprès des chefs d'entreprise, en particulier des plus petites d'entre elles, pour répondre à leurs inquiétudes

Je veux leur dire que nous travaillons avec la Fédération bancaire française et l'ensemble des banques pour que les taux d'intérêt qui pourront s'appliquer au-delà d'un an pour les extensions de prêts garantis par l'État, extensions qui sont possibles jusqu'à cinq ans, soient les plus faibles possible. Je souhaite pouvoir donner des indications précises au sujet de ces taux d'intérêt dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans quelques semaines, pour apporter de la visibilité à tous ces chefs d'entreprise. Vous avez consenti un prêt garanti par l'État (PGE) pour une

elles. Restent les autres entreprises, à savoir les PME plus importantes qui, elles, ont besoin de fonds propres. Nous travaillons à un dispositif qui permettra de compléter les prêts garantis par l'État par des instruments de quasi-fonds propres,

sera accordée à chaque entreprise qui emploie en CDI ou en CDD de plus de trois mois un jeune de moins de 25 ans payé jusqu'à 1,6 SMIC. Ce dispositif, annoncé par le Président de la République lors de son intervention du 14 juillet, sera accessible dès la fin du mois de juillet.

La troisième et dernière mesure vise les 300 000 parcours d'insertion qui seront créés pour permettre au plus grand nombre, en particulier aux jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, de trouver une solution dès le mois de septembre, que ce soit un emploi ou une formation. Ces dispositions destinées à soutenir l'emploi des jeunes font partie de ce grand plan de relance qui sera précisé, je vous l'ai dit, d'ici à la fin de l'été, et dont le Premier ministre a dévoilé les grandes orientations.

de notre pays la première économie décarbonée en Europe. La compétitivité passe bien entendu par la baisse des impôts qui pèsent encore sur nos entreprises. Depuis trente

Moi, comme élu de l'Eure, vous comme élus territoriaux, nous avons tous vu ces entreprises qui ferment, ces industries qui ne sont plus compétitives, ces ouvriers qui sont sacrifiés, ces ingénieurs qui ne trouvent plus d'emploi, parce que nous n'avons pas pris les mesures nécessaires pour engager la reconquête industrielle française.

la reconquête industrielle française est à portée de main et de volonté, mais encore faut-il que nous ayons le courage de prendre les bonnes décisions,

Encore faut-il aussi que nous ayons l'humilité de reconnaître que, en matière de fiscalité, il nous reste du chemin à faire. On ne peut pas demander à un industriel d'investir en France si les impôts de production qu'il y paie sont cinq fois plus élevés que ceux qu'il devrait acquitter s'il s'installait en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Vous connaissez le combat que je livre depuis des années sur les impôts de production.

ils obligent une entreprise à payer des impôts avant même de faire des bénéfices. Ils sont destructeurs d'emplois et pèsent sur l'attractivité de notre pays.

puisque notre objectif est d'accélérer la relocalisation industrielle en France. Nous souhaitons privilégier une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). J'ai eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises avec les régions. Dès demain, j'en discuterai de nouveau avec le président de l'Association des régions de France, Renaud Muselier. Je veux être très clair pour lever toute inquiétude : il n'est pas question que les régions paient cette baisse d'impôts. Alors, comment faire ? Il y aura donc une compensation

Elle est la condition indispensable pour une croissance durable de notre économie. Je ne crois évidemment pas à la décroissance qui conduirait tout droit à l'appauvrissement des Français et à un déclassement politique et économique inéluctable de notre pays.

C'est maintenant que notre souveraineté en matière de production d'hydrogène se joue, par exemple : soit nous investissons dès maintenant pour avoir très rapidement des entreprises capables de produire des réservoirs ou des piles à combustible,

Investir plusieurs milliards d'euros dans l'hydrogène est la meilleure façon de garantir la souveraineté politique de notre pays. Cela suppose effectivement que nous ayons une électricité décarbonée à disposition, cher Jean Bizet, celle qui nous est fournie par les centrales nucléaires. Vous le savez, je continue à croire à la pertinence de l'énergie nucléaire pour notre pays. Autre exemple de décarbonation, celle qui portera sur des projets très concrets, comme les batteries électriques, les projets de stockage des énergies renouvelables, celle qui passera par un grand plan de rénovation thermique des bâtiments.

les bonnes décisions pour la relance, non seulement nous arriverons à redresser notre économie, mais nous pourrons profiter de cette crise pour avoir, au bout du compte, une économie plus solidaire et plus respectueuse de l'environnement. Comment

finances rectificative, nous commençons à dévoiler les divers éléments de financement des plans de relance et de soutien à un certain nombre de secteurs, avant que le projet de loi de finances pour 2021 nous permette de formaliser et d'assurer le financement de toutes les mesures de relance.

étendu dans le cadre du plan Tourisme, qui a profité à plus de 1,7 million d'entreprises pour un total de plus de 3,5 millions de versements, soit près de 4 milliards d'euros engagés pour accompagner les TPE et les PME. Aujourd'hui, nous allons plus loin en injectant 500 millions d'euros supplémentaires à cette fin.

Nous voulons également aller plus loin en matière de soutien aux entreprises. Bruno Le Maire l'a dit, nous avons préparé un plan d'exonération des cotisations sociales au bénéfice des entreprises,

Les entreprises ayant des activités connexes de ces secteurs pourront bénéficier d'exonérations, dès lors qu'elles auront perdu, sur la même période, une part importante de leur chiffre d'affaires. Le travail conduit avec l'Assemblée nationale nous a permis d'élargir ce dispositif aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux non-salariés agricoles, qui pourront désormais bénéficier d'une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020, lorsqu'ils ont connu une perte d'au moins 50 Ce travail parlementaire nous a aussi permis de faciliter les plans d'apurement : les travailleurs indépendants pourront désormais les enclencher sur proposition des organismes de recouvrement. Au-delà de ces initiatives à caractère sectoriel, je tiens à souligner que nous souhaitons créer un filet de protection pour l'ensemble des entreprises. Ainsi, les entreprises de moins de cinquante salariés, qui ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur la période pourront bénéficier au cas par cas de remises de cotisations pouvant aller jusqu'à 50 % du total des cotisations dues. Comme l'a indiqué le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Le deuxième point sur lequel je souhaite m'arrêter concerne le soutien que nous voulons apporter aux territoires. Nous avons entendu les difficultés rencontrées par les collectivités locales, comme celles que connaissent l'État ou les organismes de sécurité sociale. Nous sommes convaincus de la nécessité de les accompagner et de garantir leurs ressources. Ainsi, les communes et les intercommunalités, particulièrement mobilisées pendant cette crise, qui subissent une forte altération de leurs ressources, verront ces ressources garanties. Je fais ici référence au versement mobilité, aux droits de mutation à titre onéreux

Par ailleurs, le débat à l'Assemblée nationale nous a permis de modifier la durée de remboursement des avances de DMTO en la portant à trois ans pour un montant prévisionnel qui s'élève à 2,7 milliards d'euros.

Nous avons aussi proposé à l'Assemblée nationale- elle l'a accepté -un fonds de soutien particulier à hauteur de 8 millions d'euros pour les collectivités qui profitent d'un système de financement additionnel. Je pense notamment à la Corse. Enfin, nous

à titre exceptionnel. Comme l'a dit le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ce texte prévoit nombre de dispositions permettant d'améliorer le soutien à l'économie et aux entreprises.

Les efforts que nous consentons et les dispositions que nous vous proposons sont importants. Ils permettront d'accompagner l'économie et nos concitoyens.

nous avions indiqué que le scénario de croissance était très optimiste et qu'il y avait sans doute besoin d'amplifier les mesures de soutien à l'économie. Sur ce point- nous allons y revenir tout au long des débats -, le compte n'y est pas. Il faudra des mesures de relance, dont Bruno Le Maire nous a d'ailleurs d'ores et déjà parlé. La crise est bien là, et nous devons évidemment tous être au rendez-vous pour sauver notre économie. Comme nous le savons, les chiffres sont catastrophiques : un recul de plus de 11 % du PIB, qui n'a pas de précédent depuis 1944. Malheureusement, les principales organisations internationales placent la France parmi les pays qui devraient connaître le plus fort recul de leur PIB sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Si la chute du PIB devrait être particulièrement marquée en France, les derniers développements conjoncturels suggèrent qu'elle pourrait être un peu moins forte que prévu, sous réserve bien sûr que l'épidémie ne redémarre pas.

prévision de croissance gouvernementale implique désormais que le rattrapage soit quasiment achevé, ce qui est clairement pessimiste. L'Insee anticipe, pour sa part, un recul de 9 % du PIB.

Mais il faut aussi être prudent : une nouvelle vague épidémique, qui s'accompagnerait de mesures de confinement même partielles, risquerait de provoquer une rechute de l'activité. Venons-en maintenant aux mesures figurant dans ce troisième projet de loi

Parmi les différentes composantes du plan de soutien, les mesures ayant une incidence sur le solde public connaissent une hausse de 15,5 milliards d'euros, principalement due au chômage partiel, aux exonérations de charges et aux plans de soutien sectoriels. S'y ajoutent les mesures qui n'ont pas d'effet immédiat sur le déficit public : elles sont en augmentation de 19,5 milliards d'euros. Je pense, notamment, aux reports des échéances fiscales et sociales pour plus de 7 milliards d'euros. Par comparaison avec les autres économies avancées, le plan de soutien français continue de présenter un caractère singulier, la France mobilisant moins les mesures qui ont un impact sur le déficit public, alors qu'il s'agit pourtant de dispositions pouvant apporter un soutien plus direct à l'économie. Ce différentiel paraît d'autant plus paradoxal que la France est l'un des pays où la chute du PIB est parmi les plus fortes. Cette stratégie s'explique tout d'abord par les moindres marges de manoeuvre dont dispose la France sur le plan budgétaire.

Quoi qu'il en soit, la révision à la baisse de la croissance et le redimensionnement du plan de soutien conduisent mécaniquement à une nouvelle dégradation de la trajectoire budgétaire : un déficit de 11,5 % du PIB en 2020, une nouvelle hausse de l'endettement qui atteindrait 120,9 % du PIB. Fort heureusement, il n'y aurait pas à ce stade de renchérissement des taux d'intérêt, ce qui nous laisse une certaine marge de manoeuvre. Concernant l'État, son déficit budgétaire passe

financement de l'État sont désormais colossaux : cette année, nous allons devoir emprunter 363,5 milliards d'euros sur les marchés. La situation de l'État est véritablement hors-norme : les recettes nettes diminuées des prélèvements sur recettes sont 2,2 fois inférieures aux dépenses nettes. Ainsi, le budget général connaît un déficit supérieur au montant de ses recettes et égal à 55 % de ses dépenses.

et à 2,2 milliards d'euros pour le secteur du tourisme. Les sommes annoncées par le Gouvernement incluent aussi bien des mécanismes de prêts ou des dispositifs déjà existants.

pour ma part, dès le 16 juin, un ensemble de mesures calibrées, de façon à maximiser l'effet d'entraînement sur l'activité pour un montant global de 40 milliards d'euros, soit 2 points de PIB. Le Conseil d'analyse économique suggérait 50 milliards d'euros. Malgré le fameux

En résumé, messieurs les ministres, nous ne sommes pas en désaccord avec vos mesures d'urgence et de soutien. Ce texte ne nous pose pas de difficultés, même si nous souhaitons l'améliorer.

que ces différentes mesures soient prises dès maintenant. Elles présentent également un caractère temporaire, un effet booster, pour ne pas augmenter le déficit structurel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission des finances propose d'adopter ce troisième PLFR

avant un troisième PLFR qui serait, je le pensais, celui des arbitrages politiques. J'avais alors interrogé le Gouvernement

depuis longtemps, ne semblaient pas avoir trouvé véritablement de réponse. Aujourd'hui, le temps est venu d'examiner ce texte tant attendu, mais, malheureusement, nombre de mes questions restent sans réponse ! Tout d'abord, nous sommes encore suspendus aux résultats des négociations sur les perspectives financières pluriannuelles et sur le fonds de relance européen. Les discussions vont reprendre demain. L'accord franco-allemand de mai dernier et les propositions de la Commission européenne vont dans le bon sens, encore faut-il clarifier certaines zones d'ombre- je pense notamment aux financements

un ajustement budgétaire qu'il faut bien qualifier « d'attente », du fait notamment de cette absence d'accord européen, et d'une ampleur limitée au regard du soutien dont notre économie a besoin. Les crédits nouveaux sur le budget général, soit 13,8 milliards d'euros, portent pour l'essentiel sur la mission « Plan d'urgence », entérinant notamment le coût très élevé- 31 milliards d'euros au total -du dispositif de soutien au chômage partiel, certes indispensable, mais qui nécessitera un contrôle

du fonds de solidarité pour les entreprises et des exonérations de charges, mais l'essentiel du soutien provient de simples mesures de trésorerie. Les garanties pour les entreprises avaient déjà été entérinées par le premier PLFR, avec un plafond de 300 milliards d'euros, dont chacun espère bien sûr qu'il n'aura pas lieu Tout cela est donc limité, même si le Premier ministre vient de nous annoncer un plan de relance de 100 milliards d'euros et le ministre de l'économie, des finances et de la relance, aujourd'hui même, une baisse des impôts de production de 20 milliards d'euros. Quoi qu'il en soit, les engagements pour l'avenir s'accumulent Ce collectif budgétaire était également attendu pour prendre en compte la situation des collectivités territoriales dont les recettes- versement transport, droits de mutation, taxe de séjour, octroi de mer -sont touchées par la crise. -sont touchées par la crise. Or les collectivités doivent faire face à de nouvelles charges : là encore, les propositions du Gouvernement déçoivent, avec un plan limité à 4,5 milliards d'euros, dont la moitié correspond à des avances remboursables. Nous nous reverrons donc à l'automne pour débattre de nouvelles mesures. Mais il y a urgence, car la France va connaître cette année une récession sans précédent de 11 % du PIB, selon les estimations gouvernementales, supérieure à celle de nombre de ses partenaires européens, notamment de l'Allemagne qui a pourtant décidé très rapidement d'un plan de relance bien plus massif. Il n'y a guère que le Royaume-Uni, soumis à la double peine du Brexit et du covid, qui fasse plus mal que nous Cette récession sera d'autant plus forte que nous tarderons à mettre en oeuvre les mesures de soutien nécessaires. Il y a urgence, car il s'agit non seulement de points de croissance, mais aussi des conséquences sociales : le dispositif de chômage partiel n'a apporté qu'une réponse temporaire les plans sociaux et les licenciements économiques pourraient s'enchaîner dans les mois à venir, avec des conséquences sur nos territoires. D'ores et déjà, de grandes entreprises annoncent des suppressions d'emplois : 15 000 chez Airbus, dont un tiers en France, 7 580 chez Air France d'ici à la fin de l'année 2022, 4 600 chez Renault, 1 900 chez Conforama, dont le siège est

soutenir des entreprises viables, privilégier la recherche et l'investissement, prendre en compte la responsabilité sociale et environnementale. La puissance publique dispose aujourd'hui de leviers de changement inédits et d'une opportunité historique de transformer notre économie pour le bénéfice des générations futures. À cet égard, nous cherchons encore les indices de cette transformation : conditionner une prise de participation de l'État à des engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre à travers la simple publication d'un rapport annuel, sans autre conséquence, n'est clairement pas à la hauteur des enjeux Enfin, il faudra malgré tout rester attentifs à nos finances publiques, afin de fixer un cap un tant soit peu cohérent : nous en discuterons dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques. Après des années d'application du pacte de stabilité, la crise a fait exploser tous nos repères : les déficits et la dette publique s'envolent à des niveaux que personne n'aurait pu imaginer il y a seulement quelques mois. Le Gouvernement évoque le « cantonnement » de la dette, comme si cette procédure comptable pouvait la faire disparaître ... Absolument ! ... tout en refusant de faire participer les contribuables les plus aisés à la solidarité nationale. Quand le temps de l'urgence sera passé, il nous faudra faire les comptes ... Oui ! ... et justifier la dépense publique auprès des contribuables qui seront appelés à l'assumer ! Très bien

Les indicateurs de santé publique, tout d'abord, font état d'une remontée des hospitalisations et des cas de contamination par le covid-19. Les indicateurs économiques, ensuite, évoquent une récession de 11 % pour 2020.

Les indicateurs de cohésion sociale sont également des alertes sérieuses puisqu'ils montrent que le nombre de demandeurs d'emploi et des allocataires du revenu de solidarité active explose. Il faudra bientôt y ajouter les travailleurs saisonniers, affectés par la baisse de la fréquentation touristique, et l'arrivée au mois de septembre de 800 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Si l'on y adjoint la très faible participation lors des élections municipales, nous nous trouvons face à un parfait cocktail explosif d'une crise de sens et d'unité populaire, donc d'une crise politique sur fond de confinement de la démocratie

social ni d'un tournant écologique. Il ne sera pas question non plus de revenir sur les cadeaux fiscaux aux plus riches, mais il faudra en revanche travailler plus et faire payer encore une fois les salariés et les retraités de ce pays vrai ! Ce que révèle surtout cette intervention présidentielle, par ailleurs on ne peut plus paternaliste, c'est que le Gouvernement continue de privilégier la communication politique du « en même temps » au détriment de l'action politique. Avec ce troisième PLFR et les annonces dites de soutien ou de relance,

niveau, pour collecter plus de 160 milliards d'euros d'ici à 2042 ! Cela dit, il aura fallu attendre un troisième texte financier pour voir un plan de soutien aux collectivités annoncé en grande pompe. Mais si l'intention est bien là, le compte n'y est pas ! Le Gouvernement a demandé au député Jean-René Cazeneuve-ce n'est pas un député communiste ! -de faire le point sur les pertes financières des collectivités. Si nous reprenons ses premiers résultats, notre collègue chiffre la perte à 7,5 milliards d'euros pour 2020 : 3,2 milliards d'euros pour le bloc communal, 3,4 milliards d'euros pour les départements et 0,9 milliard d'euros pour les régions.

par des entreprises pourtant soutenues par l'État, et qui aujourd'hui se permettent d'organiser des plans sociaux et des délocalisations en toute impunité ? Quant aux régions, ne cherchez pas, mes chers collègues, il n'y a rien La réactivité et l'inventivité des collectivités territoriales ont été sans commune mesure. Elles ont permis de tenir la barre à travers la tempête du covid-19. Malgré les signaux contradictoires reçus d'en haut, voire parfois l'absence de signaux, les collectivités locales ont prouvé la solidité de l'organisation territoriale française,

la solidité financière. La confiance des Françaises et des Français appelait un nouveau chemin d'égalité sociale et territoriale. Ce projet de loi de finances rectificative n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas. Pour les élus du groupe

le sauvetage de notre économie est loin d'être terminé que la relance doit déjà commencer. C'est une nécessité impérieuse pour sauvegarder nos entreprises et l'emploi, et tracer des perspectives d'avenir. Telle devra être l'ambition de ce troisième projet de loi de finances rectificative qui nous est présenté et dont nous entamons aujourd'hui l'examen. La montée en puissance des dispositifs doit se poursuivre. Si la propagation du virus semble pour le moment avoir été maîtrisée, même si nous devons redoubler de prudence, la crise économique, quant à elle, ne fait malheureusement que commencer. S'il faut se prémunir contre une deuxième vague épidémique à l'automne, il faut aussi craindre une vague de difficultés économiques, déjà perceptible sur nos territoires. C'est C'est pourquoi nous devons continuer à déployer des mesures pour soutenir nos entreprises et l'emploi. C'est l'aspect défensif de la politique qui est menée depuis le mois de mars. Il est essentiel, car il a permis à notre économie de tenir. Sans entreprises, pas de reprise

la relance en plus de prévoir le sauvetage. Ce troisième volet du plan de sauvetage de l'économie vise à amplifier la réponse globale. Je pense, notamment, à l'abondement supplémentaire au fonds de solidarité pour les PME, les TPE et les indépendants ou aux compensations de cotisations sociales pour les entreprises les plus touchées. Au-delà de ces mesures, d'autres plus spécifiques complètent utilement les dispositifs de soutien pour les secteurs les plus exposés à cette crise : automobile, aéronautique.

Je me réjouis également que le Gouvernement ait fait le choix de privilégier une action publique au plus près du terrain et des collectivités. C'est notamment le cas avec la possibilité laissée au bloc communal de procéder à des dégrèvements exceptionnels de cotisation les plus touchées, ainsi qu'à des exonérations de taxe de séjour en 2020. Il s'agit là de faire confiance aux acteurs de terrain qui connaissent le mieux les difficultés et les réalités locales. Néanmoins, les délais sont trop contraints. Il n'est pas sérieux d'imaginer que les EPCI, à peine installés, ou les communes pourront prendre de telles décisions avant le 31 juillet, soit quelques jours à peine après la promulgation de la loi.

Le plan de soutien, dont le montant global s'élève à 4,5 milliards d'euros, va bien évidemment dans le bon sens. Mais je crois que nous devons encore en accentuer l'ambition. Je suis certain que le Sénat y sera particulièrement vigilant. Il y va de l'intérêt général de la Nation et de sa cohésion. Je pense, notamment, à la dotation instituée par l'article 5, qui vise à compenser les pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l'épidémie.

et à titre de comparaison, dès le début de la crise financière, nous avons voté des mesures de soutien aux petites entreprises par le biais du fonds de solidarité, avec un minimum de 1 500 euros.

et à la Banque européenne d'investissement, pour des montants respectifs de 4,4 milliards et de 4,7 milliards d'euros. Toutes ces mesures sont nécessaires pour préserver

les réponses apportées par l'État dans le cadre des deux premières lois de finances rectificatives ont été immédiates et massives. Certes, les mesures étaient coûteuses, mais elles étaient absolument nécessaires au regard de la déflagration économique, financière et sociale provoquée par la pandémie de covid-19. Il s'agissait d'éviter l'effondrement de nos entreprises et ses conséquences sociales, de sauver notre tissu économique, les emplois dans les territoires, de protéger les plus fragiles, au moment où l'économie de notre pays et celle de nos voisins étaient à l'arrêt. Avec ce troisième projet de loi de finances rectificative, le coût budgétaire des grandes mesures de soutien à l'économie et à l'emploi sera porté à environ 50 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent près de 70 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales,

mais pouvait-il en être autrement compte tenu de l'urgence qu'il y avait à soutenir nos entreprises, leurs salariés et, au-delà, les plus fragiles de nos concitoyens ? Désormais, un deuxième rendez-vous, tout aussi important, nous attend : celui de la relance. Nous devons absolument le réussir ! Relancer la machine économique tout en saisissant les opportunités qui nous sont données de transformer durablement nos modes de production, de reconquérir notre souveraineté dans des domaines stratégiques, de faire de la transition écologique un moteur de développement des territoires et de la justice sociale le ferment de la cohésion nationale, telle doit être notre feuille de route. Il s'agit d'opportunités parfois exigeantes, mais elles sont réellement cruciales pour l'avenir de notre société. Ce PLFR amorce ce virage en soutenant les secteurs les plus durement touchés- tourisme, culture, automobile, aéronautique, nouvelles technologies -, tout en s'inscrivant dans la perspective de la transition écologique. À ce titre, nous saluons l'ajout de l'article 19 conditionnant les prises de participation de l'Agence des participations de l'État au sein du capital des grandes entreprises à la souscription d'engagements en matière de transition écologique. Au-delà de l'inquiétude que suscite le dévissage de nos finances publiques, c'est bien la multiplication des destructions d'emplois et la perspective de milliers de jeunes sans débouchés immédiats qui doivent nous alerter. On nous annonce pas moins de 800 000 suppressions d'emplois d'ici à la fin de l'année, alors que, dans le même temps, arriveront tout d'un coup plus de 700 000 jeunes sur un marché du travail fragilisé. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons accueilli favorablement les différentes annonces qui ont été faites dans ce domaine, qu'il s'agisse des primes pour l'emploi d'un apprenti ou de la réduction du coût d'embauche des jeunes.

Quoi qu'il en soit, ce PLFR va dans le bon sens et nous approuvons l'exonération de cotisations et de contributions sociales et patronales prévue à l'article 18. Associé à un crédit de cotisations, il s'agit là d'un dispositif inédit qui bénéficiera automatiquement à un grand nombre de secteurs de l'économie : l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, le sport, la culture, ou encore le transport aérien. L'article 18, dont le champ d'application a été opportunément étendu, comporte en outre un filet de sécurité pour toutes les entreprises, indépendamment de leur secteur d'activité. Cela nous paraît aussi bienvenu. Bien sûr, sur tous ces sujets, la copie gouvernementale reste perfectible et la commission des finances, comme mon groupe, proposera des amendements visant à l'améliorer. tout au long de cette crise, le besoin de remettre le local au centre de notre modèle s'est manifesté avec force à l'échelle du pays.

À ce titre, je regrette que ce collectif budgétaire ne prenne pas suffisamment en compte la situation des départements. Ces derniers pourraient pourtant demain apporter leur pierre à la dynamique économique des territoires. L'avance proposée pour compenser les pertes de recettes des DMTO de 2,7 milliards d'euros est certes nécessaire, mais cette mesure doit être complétée. Nous proposerons par conséquent des améliorations. En revanche, le soutien apporté, à hauteur de 1,7 milliard d'euros, en faveur de l'investissement du bloc communal nous paraît décisif. C'est l'une des vertus de ce budget rectificatif que de prévoir, là encore de façon inédite, une compensation intégrale des pertes de recettes fiscales et domaniales des communes et intercommunalités. En ouvrant par ailleurs 1 milliard d'euros de crédits supplémentaires de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), ce budget préfigure la relance à venir dans les territoires autour de la transition écologique, de la résilience sanitaire, mais également, et c'est important, de la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. Sur ce sujet, monsieur le ministre, il me semblerait opportun que ces crédits soient, pour la moitié au moins, fléchés vers les préfets de département. Ce serait un beau message adressé à l'échelon départemental, à l'échelon local qui, tout au long de la crise sanitaire, a su répondre dans la proximité, avec agilité et efficacité aux besoins des habitants. Enfin, le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en année pour toutes les collectivités serait de nature à accélérer l'investissement local. Nous défendrons un amendement en ce sens. Pour conclure, sachez, monsieur le ministre, que dans un esprit toujours positif les membres du groupe Union Centriste auront à coeur, au cours de ces trois prochains jours, d'enrichir ce texte qui va dans le bon sens, et qu'ils soutiendront dans leur grande majorité. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs en mars dernier, le Président de la République annonçait une France « en guerre ». Aujourd'hui, l'ennemi invisible est moins prégnant, mais toujours menaçant, tandis qu'une bataille reste à gagner : celle de l'emploi. Elle en cache d'autres : la bataille de la justice sociale et la bataille des territoires. Le Premier ministre l'a rappelé ce matin, la crise de la covid a accentué certaines fractures au sein de notre modèle économique et social. et social. L'urgence sanitaire demeure, et une deuxième vague est possible dans notre pays. C'est dans ce contexte sanitaire incertain qu'il nous faut relancer l'économie dans les prochains mois. L'équation n'est pas facile : l'incertitude affecte l'indice de confiance du côté tant des ménages que des entreprises. Aussi, le succès de la relance sera conditionné à la à la capacité de l'exécutif de dynamiser en même temps l'emploi, l'investissement et la consommation. À ce stade, les « airbags » jouent leur rôle. Toutes les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement aident notre économie à surmonter le choc du confinement, du moins à court terme. Regardons le recours au chômage partiel. Il a permis de protéger les ménages en limitant la chute de leurs revenus à 3,2 % pendant le confinement, alors qu'au même moment le revenu national baissait de près d'un tiers, selon l'Insee. Le soutien au pouvoir d'achat, au travers du dispositif d'activité partielle, a ainsi permis à la consommation des ménages de rebondir plus fortement que prévu : en juin, l'activité économique a déjà comblé près des trois cinquièmes de l'écart qui la séparait, au pic du confinement, de son niveau d'avant la crise.

Quant aux outils de soutien à la liquidité des entreprises, ils ont également fait leurs preuves. Avec 105 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, la France est le pays européen dans lequel cette forme de soutien a été la plus fortement mobilisée Ce volume important a certainement contribué à repousser le risque d'une grande vague de faillites, en permettant aux entreprises d'étaler l'incidence du confinement. Cependant, comment contenir les plans sociaux qui pourraient se présenter dès l'automne ? Le Président de la République l'a plusieurs fois déclaré : « La rentrée sera difficile. En effet, en dépit de ces mesures de soutien, les pertes de revenus des entreprises restent très importantes : 54 milliards d'euros entre les mois de mars et de juillet. Une demande insuffisante, je l'ai dit, et la contraction de l'économie mondiale vont durablement peser sur l'activité. Soyons réalistes : pour faire face à cette récession sans précédent et afin que les difficultés conjoncturelles ne se transforment pas en crise durable, la France devra consentir un effort public soutenu soutenu et encore plus important. C'est l'objet de ce troisième projet de loi de finances rectificative, qui, tout en assurant la continuité des mesures précédentes, a le mérite de cibler les secteurs les plus touchés. Comme on le sait, les conséquences du confinement sont dramatiques sur l'aéronautique, le tourisme et la culture. Par rapport à d'autres pays européens, nous sommes là face à une vraie difficulté, car les avantages comparatifs de la France se situent dans des secteurs structurellement plus exposés la fermeture des économies mondiales. Alors, comme l'a souligné avec pertinence la commission des finances, ce soutien sera-t-il suffisant au regard des enjeux que représentent ces secteurs, poids est fondamental pour notre économie et l'équilibre de nos territoires ? La dégringolade, au fil des budgets rectificatifs, de la prévision de croissance pour 2020 témoigne de la spécificité française. Alors qu'elle

une hausse massive du déficit conjoncturel par rapport aux projections de la loi de finances initiale, soit une baisse de 7,1 points de PIB, une dette publique qui pourrait atteindre les 121 % d'ici à la fin de l'année. Ces chiffres nous auraient horrifiés il y a seulement quelques mois. Mais, partout au sein de la zone euro, la ligne rouge a été franchie dans un contexte- je le rappelle -où la règle européenne qui fixe le niveau d'endettement à 60 % du PIB maximum est devenue obsolète. Le risque d'effondrement économique a pris l'avantage sur la question de la dette et la sacro-sainte orthodoxie budgétaire. Pouvons-nous faire autrement ? Je ne le crois pas et mon groupe vous soutient, monsieur le ministre, dans cette direction, pourvu pourvu qu'elle soit provisoire. Mais dans cette entreprise de remobilisation économique, nous avons besoin de tous les leviers.

quant à la compensation de leurs recettes fiscales, car nos collectivités locales vont jouer un rôle fort d'amortisseur social dans les mois qui viennent, ce qui implique le maintien de leurs moyens budgétaires. Monsieur le ministre, vous le savez, les régions s'inquiètent du projet de baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, même si l'on peut comprendre le principe d'un allégement des impôts de production. Mes chers collègues, nous examinons ce projet de loi de finances rectificative alors que se profile déjà un nouveau plan de relance annoncé par le Président de la République, et relayé par le Premier ministre. Doté d'au moins 100 milliards d'euros, un programme de cette ampleur nous permet de mieux envisager l'avenir et de rendre de l'espoir à tous les acteurs économiques. Je pense en particulier aux jeunes : ils doivent entendre autre chose que la promesse d'un horizon de dettes qui s'amoncellent. Comme vous le savez, ils seront près de 700 000 en septembre à postuler à un emploi ! Le dispositif exceptionnel d'exonération des charges jusqu'à 1,6 SMIC annoncé me semble tout à fait intéressant et essentiel à l'insertion de la jeunesse qui entre sur un marché du travail en pleine récession. Cependant, peut-être pourrons-nous aller un peu au-delà de ce seuil, de façon à toucher également les diplômés de l'enseignement supérieur. Nous en reparlerons ... Pour finir, je Pour finir, je rappellerai l'entier soutien du RDSE au plan de relance européen Next Generation EU, pas seulement parce qu'il pourrait profiter à la France à hauteur de 40 milliards d'euros, mais parce qu'il concrétise un effort de solidarité, au travers d'une forme de mutualisation des dettes, nécessaire nécessaire à la cohésion de l'Union européenne. Il reste à souhaiter que tous les États membres en soient convaincus pour que ce plan soit rapidement mis sur pied ; nous le souhaitons ardemment. En attendant, mes chers collègues, nous examinerons avec bienveillance

J'ignore si tel est le cas. Les formules de Paul Valéry sont parfois mystérieuses ... En tout cas, tout doit recommencer après une interruption. Les signaux, pas seulement sanitaires, sont contradictoires de ce point de vue. On annonce une contraction inédite, inédite, à moins 11 %, mais aussi des capacités de rebond, soulignées par la Commission européenne, l'Insee, ou encore la Banque de France. Nous sommes donc à la croisée des chemins.

en particulier grâce aux primes exceptionnelles à l'embauche des apprentis ; il accompagne les collectivités territoriales en prévoyant jusqu'à 4,5 milliards d'euros

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà voté deux projets de loi de finances rectificative et plus de 460 milliards d'euros de mesures sectorielles depuis le début de l'épidémie.

Les prévisions de croissance pour 2020 annoncent une chute de 11 % du PIB et une perte de 1 million d'emplois, et nous en sommes toujours à discuter de 43 milliards d'euros supplémentaires. En Allemagne, le gouvernement fédéral a injecté près de 130 milliards d'euros, soit une ambition trois fois supérieure à la nôtre Je rappelle tout de même que le présent projet de loi fait exploser notre déficit de 11,4 % et porte notre dette publique à 120 % du PIB. C'est un poids colossal que nous devrons assumer et que nous faisons déjà supporter par les générations futures. Certes, cette crise économique est due à la crise du coronavirus, que coronavirus, que vous n'avez pas su gérer, mais elle aussi le résultat de vos choix politiques et économiques des dernières décennies. Avec 8 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, votre projet manque à l'évidence d'ambition pour soutenir les TPE et PME. On ne peut pas cantonner les exonérations de charges aux entreprises contraintes à une fermeture administrative. Il faut élargir le périmètre aux sous-traitants et aux fournisseurs pendant la durée nécessaire à la reprise d'une activité normale, c'est-à-dire identique aux mois précédents, compte ! À la rentrée, le chômage des jeunes va exploser : 50 000 apprentis sont menacés d'ici au 1 septembre, et 800 000 jeunes arriveront sur le marché du travail à la même période. La baisse des taxes pour l'embauche des jeunes, si elle se produit, ne suffira pas à absorber un tel choc. Il est temps de revoir l'efficacité décisionnelle de nos politiques en consacrant le principe de subsidiarité, en supprimant les échelons de décision inutiles, comme les agences régionales de santé (ARS), qui ont fait preuve de leur inefficacité, régionaux (CESER), et certaines intercommunalités qui coûtent tant et rapportent si peu. Il faut s'affranchir du carcan européen, qui a brillé par son inaction durant la crise sanitaire. En parallèle, nous dégagerons des moyens financiers, nous baisserons la dépense publique inutile et nous pourrons redonner une autonomie financière aux communes qui se sont tant battues, et souvent seules. Par ailleurs, le soutien aux entreprises par le recours au chômage partiel et les 31 milliards d'euros qui sont prévus est une bonne chose, car protéger les entreprises, c'est protéger les salariés. Cependant, le parquet de Paris a annoncé qu'il enquêtait sur des escroqueries massives. Votre ministère doit impérativement border le dispositif pour éviter la fraude, monsieur le ministre. Nous sommes en récession en raison de votre impréparation et de votre incompétence durant la crise du coronavirus. Ce ne sont pas le discours de politique générale de ce matin, qui ressemblait à un réquisitoire contre la politique appliquée-

Les textes devaient s'enchaîner pour tenter de contenir les effets de la crise, qui s'annonce très profonde, mais, souhaitons-le, avec un rebond substantiel possible dès 2021, à la condition de prendre les bonnes décisions en temps et en heure. heure. Parmi les questions que nous devons nous poser au moment d'examiner ce texte, celle du tempo des mesures est au moins aussi importante que celle du contenu. Le Gouvernement avait qualifié les deux premiers textes « d'urgence », « de sauvegarde », et celui-ci de finances rectificative aurait pu être- rien ne vous en empêchait -, outre un plan de soutien complémentaire aux secteurs les plus en difficulté de notre économie, le grand plan de relance annoncé en fait depuis mars, dont les mesures, si elles avaient été adoptées en juillet, auraient pu être opérationnelles à la rentrée, au moment notamment où 700 000 jeunes arriveront sur le marché du travail et où, c'est à craindre, le nombre des défaillances d'entreprises va commencer à augmenter. à augmenter. Le Gouvernement a fait un autre choix sans que nous en comprenions vraiment les raisons, sauf à considérer que le changement de Premier ministre et le remaniement ministériel ont bouleversé l'agenda. Le Parlement aurait pu travailler trois ou quatre semaines de plus avant la coupure estivale

revenir un instant sur la situation de la France d'avant et le tableau qu'en brosse généralement Bruno Le Maire. C'est aujourd'hui notre point de départ, avant la crise. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance met souvent en avant le net recul du chômage, sous les 8 %- c'est exact -, le regain d'intérêt pour l'apprentissage- exact là aussi -, la bonne tenue de l'investissement privé- exact également -, et même la bonne tenue de la consommation des ménages jusqu'en 2019- exact encore. Permettez-moi cependant de relativiser ces propos en rappelant simplement quelques chiffres. Ceux de la croissance, d'abord : 2,3 % en 2017 ; puis 1,8 % en 2018 Une belle pente descendante, avec un acquis de croissance de seulement 0,1 % pour 2020, avant la crise, ce qui est le plus mauvais chiffre depuis 2012. Ceux du déficit du budget de l'État,

viens au déficit public : 3 % du PIB en 2019. Pour la première fois depuis 2011, il est reparti à la hausse. Quant à la dette publique, elle a frôlé l'an dernier les 100 % du PIB.

Nous avons abordé la crise dans une situation économique et financière bien plus dégradée que la plupart des autres États européens. En 2019, nous étions en queue de peloton : sur 27, nous étions nous étions 23 pour la croissance et l'endettement public, 24 pour le taux de chômage, 26 pour le déficit public. Même avec un taux de chômage de 8,1 % en février dernier, seules l'Italie, l'Espagne et la Grèce faisaient moins bien que nous. Avec un taux de croissance de-0,1 % au quatrième trimestre 2019, seules l'Italie, la Finlande et la Grèce faisaient moins bien que nous. Avec 98,1 % de taux d'endettement, seuls la Belgique, le Portugal, l'Italie et la Grèce faisaient moins bien que nous.

Mais maintenant, l'incendie à éteindre est d'une tout autre ampleur et il y a urgence. Nous n'avons pas dix ans devant nous. Voilà pourquoi nous pensons que vous perdez du temps par rapport à nos grands voisins. M. Le Maire a beau nous dire que l'effort de la France est comparable à celui de l'Allemagne, notre rapporteur général démontre, dans son rapport, qu'il n'en est strictement rien.

! Pourtant, au début de la crise, le Président de la République a utilisé l'expression, probablement hasardeuse, « quoi qu'il en coûte ». Et le 14 juillet dernier, il nous a annoncé un plan de relance de 100 milliards d'euros. Mais quand et comment, nous ne le savons pas exactement. Considérant que notre économie ne peut attendre six mois de plus, mon groupe déposera des amendements sur ce texte, comme notre rapporteur général, au nom de la commission des finances, mais aussi les autres commissions, à commencer par celle des affaires économiques, économiques, qui ont travaillé, auditionné, préparé des mesures de relance. Les sénateurs Les Républicains proposeront ainsi de baisser les impôts de production, afin d'améliorer la compétitivité de nos entreprises

et par la suppression du forfait social pour les PME et les ETI. Nous proposerons également de baisser les charges sociales, pour diminuer le coût du travail et lutter contre le chômage, en soutenant l'emploi des jeunes et la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi. Nous proposerons de doper les investissements dans le capital des entreprises. La plupart d'entre elles sont aujourd'hui fragilisées et la question de leur solvabilité va être essentielle. Leurs besoins en fonds propres sont estimés entre 10 et 30 milliards d'euros par la Banque de France, un montant considérable. Les chiffres sont éloquents : l'effondrement des recettes fiscales de 66 milliards d'euros sera dû, pour moitié, à l'effondrement des bénéfices des entreprises, avec une perte estimée, pour 2020, à 32,4 milliards d'euros de recettes d'impôt sur les sociétés. La chute de la consommation, avec 19,8 milliards de baisse des recettes de TVA, ne vient qu'en second. Les revenus des ménages n'ont diminué, pour leur part, si j'ose dire, que de 6 milliards d'euros. Nous proposerons aussi de renforcer le soutien à certains secteurs, comme les transports et le logement, des secteurs clés dont dépend aussi le bon fonctionnement de notre économie.

insuffisantes. Notre rapporteur général vous proposera d'aller plus loin, afin que la région capitale, où la qualité des transports en commun est vitale pour nos entreprises et où les besoins sont- c'est le moins que l'on puisse dire -considérables, ne soit pas laissée pour compte. Quant au logement, si l'accent est mis sur la rénovation thermique de l'existant- sujet certes important -, nous n'avons pas vraiment le sentiment que tout soit fait pour soutenir la construction neuve. sont, là aussi, réels. Les emplois concernés sont non délocalisables et la chute du nombre de logements construits, tant dans le parc privé que dans le logement social, ne pourra qu'alimenter la fournaise des prix, que nous n'arrivons toujours pas à enrayer.

Nous soutiendrons également des mesures favorisant la transition énergétique, notre conviction étant que le rebond passera aussi par la croissance écologique et non par la décroissance verte, comme l'a très justement souligné M. le Premier ministre. Enfin, nous proposerons de soutenir la consommation, qui a fortement chuté, au travers de mesures visant à libérer l'épargne des Français, qui s'est accumulée pendant le confinement. Les estimations varient entre 75 milliards et 100 milliards d'euros, c'est considérable la relance de la consommation des ménages dépendra aussi de la confiance des Français, qui repose sur plusieurs éléments : le maintien des filets sociaux de sécurité, mais aussi la stabilité fiscale promise par le Président de la République. De ce point de vue, nous regrettons les propos contradictoires qui sont exprimés à ce sujet au sein de votre majorité, monsieur le ministre. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pourtant réputé proche du Président de la République, a laissé entendre qu'il faudrait davantage taxer les premiers de cordée,

de son entretien du 14 juillet dernier, que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de ménages les plus aisés serait sans doute reportée ; mais reportée comment et de combien de temps ? Nul ne sait et Mme Gourault était, ce matin, à la télévision, bien en peine d'expliquer ce qu'il en est ce qu'il en est ... Nous étions opposés à la suppression de la taxe d'habitation, qui coûte très cher à l'État- 17 milliards d'euros par an -et qui va couper le lien fiscal entre,, la moitié des habitants et leur commune,

En ce qui concerne la relance verte, et pour soutenir la filière automobile, nous vous proposons d'augmenter le bonus écologique en supprimant les conditions de ressources pour l'attribution de la prime à la conversion en faveur d'un véhicule propre. Nous souhaiterions également que le bonus écologique soit élargi aux véhicules électriques ou à hydrogène d'occasion et que la prime à la conversion soit rétablie dans sa version antérieure au mois de juillet 2019. En matière de soutien à nos agriculteurs, qui ont également souffert de la crise, nous prônons la mise en place d'une aide compensant 50 % de leurs pertes d'exploitation s'ils ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires supérieure à 30 %.

Quant au soutien aux demandeurs d'emploi, nous demandons que soit abaissé de 1 000 à 500 le seuil au-delà duquel une entreprise doit offrir un congé de reclassement à ses salariés en cours de licenciement et nous souhaitons que ce mécanisme soit étendu à au moins une année. Cette mesure pourrait être utilement combinée avec le dispositif de chômage partiel de longue durée.

les doublons dans notre organisation territoriale, d'achever la décentralisation et de diminuer le nombre d'agences de l'État. Eh oui ! Malheureusement, le temps est devenu très court et nous allons devoir réformer en pleine crise. Comme François Hollande, Emmanuel Macron n'a eu de cesse de repousser les efforts à plus tard, et voilà que nous allons devoir faire ces réformes structurelles au moment où ce sera le plus difficile.

de 11 %- c'est le chiffre retenu dans ce collectif budgétaire -, cela signifie une perte de 267 milliards d'euros. Cette baisse est à comparer avec celle de 2,9 % en 2009 ; le choc de cette crise sera donc trois fois supérieur à celui de la crise de Le taux de dépenses publiques passera ainsi mécaniquement de 54 % à 63 %, un niveau jamais atteint. Pour financer tout cela, nous n'avons pas d'autre moyen, dans un premier temps, que de laisser filer le déficit

dette comme vous le voulez, monsieur le ministre, logez-la où vous voulez, mais ayons tous le courage de dire aux Français qu'il faudra bien la rembourser, qu'il faut faire les efforts nécessaires. Absolument ! Alors, disons-le collectivement, c'est le meilleur moyen d'entraîner le pays tout entier.

nous sommes amenés à examiner un texte présentant un déficit de plus de 11 % du PIB et une dette de plus de 120 % du PIB. Mes chers collègues, nous aurions tous été horrifiés, si l'on nous avait annoncé cela au mois de décembre dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances initial pour 2020 pourtant, nous en sommes là ... Je note la nature très ambivalente de ce texte, qui n'est ni pleinement un plan d'urgence ni véritablement un plan de relance.

des prêts garantis par l'État- lesquels, nous l'espérons, ne seront pas toujours appelés -, ou encore des reports de charges ... Autant de décisions qui ont des effets directs sur le budget de l'État, mais également sur les dépenses de sécurité sociale et de retraite, en raison d'exonérations non compensées par ailleurs, que de nombreux crédits sont ouverts pour traiter des conséquences de la crise sanitaire et économique que nous connaissons. Toutefois, le groupe socialiste et républicain du Sénat ne peut que déplorer le manque d'ambition de ce projet parti socialiste et ses deux groupes parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont produit un plan de relance, présenté à la presse le 9 juin dernier. Ce plan identifiait ce que nous considérons comme des manques flagrants dans l'action du Gouvernement. Nous pensons qu'il faut aller plus loin dans le soutien à certains secteurs et dans le rééquilibrage de l'économie, tant sur le volet social que sur le volet environnemental. Des quarante-cinq propositions que nous avons formulées à cette occasion,

qui nous semble d'autant plus nécessaire que le Gouvernement tarde à mettre en oeuvre un vrai plan de relance et qu'il multiplie certaines annonces contradictoires

Vous pouvez bien le nier, cela n'en demeure pas moins la stricte vérité. Comble de l'ironie, vous n'assumerez même pas ce nouvel impôt, qui interviendra à partir de 2024. Ainsi, chaque Français, y compris parmi les plus modestes, sera mis à contribution sans qu'aucune progressivité soit prévue. Nous demandons, une nouvelle fois, davantage de justice sociale et fiscale et nous vous proposerons des mesures allant dans ce sens : rétablissement de l'ISF, suppression de la, réintroduction de la taxe sur les hauts salaires, contribution exceptionnelle des encours d'assurance vie les plus élevés, renforcement de la taxe sur les transactions financières et sur les dividendes. Vous avez l'embarras du choix,

Cela permettrait d'avancer sur un chemin nouveau- non un « nouveau chemin » -socialement plus juste, alors que, aujourd'hui, en exemptant les plus riches au détriment de nos enfants et de nos petits-enfants, vous faites le choix de l'irresponsabilité du « quoi qu'il en coûte », financé par de la dette. Deuxième point : la culture, au sens le plus large du terme. Nous avons le sentiment que le Gouvernement ne prend pas véritablement la mesure de la gravité de la crise que traverse ce secteur. Nous proposerons, au lieu d'une multitude de petits amendements très spécifiques, la mise en place d'un plan global de sauvegarde et de relance de la vie culturelle dans notre pays. C'est indispensable et très complémentaire d'une politique touristique. Troisième point, qui doit absolument être musclé : la transition environnementale. Il s'agit non pas de contraindre un tissu économique en souffrance, mais de préparer l'économie de demain, en instaurant des mécanismes de fléchage des fonds et de conditionnalité de certaines aides. La majorité présidentielle a introduit, à l'Assemblée nationale, un amendement en la matière, mais nous estimons qu'il faut aller au-delà du voeu pieux et trouver un équilibre entre incitation et obligation ; ce n'est pas le cas, à ce stade.

Quatrième point : les collectivités territoriales. Nous devons garantir le niveau de ressources de celles-ci, car c'est dans les territoires, avec l'appui des élus locaux, que nous pourrons disposer des leviers les plus efficaces pour relancer les systèmes productifs locaux. En effet, les choix successifs en matière de fiscalité locale conduisent à une disparition de l'autonomie fiscale, comme en témoigne l'annonce du projet de suppression des impôts de production, comme la CVAE, perçue par les

C'est dans cette perspective que nous avons souhaité garantir leur niveau de ressources et favoriser une réflexion et l'engagement d'une action publique résolument dynamique en matière de transports urbains au sens large, mais aussi de mobilités urbaines, avec l'effort désormais incontestable en matière de circulations dites « douces J'aurais pu aborder de nombreux autres points, comme la recherche, l'enseignement supérieur, l'emploi, la lutte contre le chômage des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, ou encore l'agriculture et l'alimentation, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. mots, mes chers collègues, l'état d'esprit dans lequel nous abordons ce texte. Vous l'aurez compris, le vote du groupe socialiste et républicain dépendra du sort réservé à ses propositions. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre,

il n'y ait aucun gel, aucun report, aucune annulation de dépenses. Nous avons entendu le Président de la République indiquer que l'on allait reporter la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % restants des ménages, mais,

il était temps qu'un projet de loi de finances rectificative prévoie enfin des crédits et engagements pour nos compatriotes français de l'étranger, qui subissent de plein fouet la crise pandémique. Lorsque l'on est expatrié, on est étranger dans le pays d'accueil, et, en tant que tel, on a, à la fois, peu de droits et le devoir de respecter les règles du pays d'accueil. S'il y a des licenciements, ce sont les étrangers qui voient leurs contrats interrompus, sans indemnités ; ils doivent pourtant continuer de faire vivre leur famille. Les membres de certains couples français ont tous les deux perdu leur emploi. Ils ne veulent pas rentrer pour autant, mais il leur faut du temps pour retrouver un emploi et faire face à leurs dépenses. De plus, dans beaucoup de pays, les permis de séjour sont liés aux contrats de travail. Le plan de soutien prévoyait un dispositif de 50 millions d'euros de crédits, destiné à aider nos compatriotes les plus démunis touchés par la crise. Deux mois après l'annonce de cette aide exceptionnelle, seulement 2 700 de nos compatriotes ont pu bénéficier de cette aide, totalisant à peine 390 000 euros, soit moins de 1 % de l'enveloppe destinée à soutenir les Français de l'étranger en grande difficulté. Serait-ce parce que, finalement, ces Français résidant hors de France vont mieux ? Pas du tout, mais les critères d'attribution de ces aides sont opaques et mal connus. Ils ne font pas l'objet d'un texte réglementaire ; nul ne comprend pourquoi tant de personnes ne sont pas éligibles à ces subventions, alors qu'elles se retrouvent, brutalement, totalement démunies. Les dossiers sont étudiés par les postes diplomatiques, dont la compétence n'est pas remise en cause, mais qui n'ont pas toujours une parfaite connaissance de la situation individuelle des personnes en difficulté.

Les conseillers des Français de l'étranger nous font part de leur totale incompréhension face à l'obligation de ne verser cette aide qu'une seule fois, alors que, chacun en convient et l'annonce, la crise sera longue. En tout état de cause, cette aide est totalement sous-dimensionnée par rapport aux besoins. de toute urgence, des critères adaptés, qui tiennent compte des problèmes individuels de chacun et qui permettent de payer le loyer, la scolarité et les frais de la vie quotidienne pendant au moins six mois, quitte à ce qu'il s'agisse d'un prêt remboursable. Il faut donner la possibilité d'utiliser cette subvention, à moins qu'elle ne soit qu'un leurre ... Les Français qui ont créé de petites entreprises à l'étranger connaissent également des difficultés. M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État, avait donné quelques espérances en réponse à ma question d'actualité du 1 juillet. Il avait reconnu des lacunes concernant nos entreprises en déclarant : « Je souhaite mettre en place un volet complémentaire, à à destination des entrepreneurs, dont certains ne bénéficient pas d'aides locales ; je suis en train d'y travailler avec mes collègues de Bercy. » Or il n'y a aucun crédit ni aucune mesure pour ces entreprises dans ce Il est urgent de mettre en place un plan de soutien aux entrepreneurs français à l'étranger qui permette à ceux-ci d'obtenir le financement de six mois de trésorerie par des avances remboursables à partir de 2022. qui concerne nos établissements scolaires français à l'étranger, il a été, là encore, prévu une enveloppe de bourses supplémentaires pour faire face aux frais de scolarité, que les parents ne veulent ou ne peuvent pas régler, en particulier du fait de l'enseignement à distance. Malheureusement, les établissements scolaires n'ont pas d'autre choix que de facturer l'intégralité des écolages, déduction faite des frais n'ayant pas été supportés. Là aussi, l'information n'a pas été correctement diffusée. Les décisions d'octroi sont prises non pas sur place, par les personnes qui connaissent les situations des familles, mais à Paris, et les critères sont également totalement opaques. La plupart des dossiers sont refusés. On va encore nous dire que la totalité de l'enveloppe des bourses n'a pas été consommée, alors que beaucoup de familles ne peuvent pas payer le troisième trimestre et risquent de ne pas réinscrire leurs enfants l'année prochaine. Cela est susceptible de mettre en grande difficulté les établissements eux-mêmes. Quand on compare les centaines de milliards d'euros distribués en France et en outre-mer aux 220 millions d'euros qui ne seront même pas totalement distribués à l'étranger, on a le droit de s'interroger. En France, c'est « quoi qu'il en coûte ». Nous aimerions qu'il en soit ainsi pour les Français résidant à l'étranger. Il serait regrettable que l'on soit obligé de rapatrier ceux qui n'auront pas réussi à passer la vague, simplement parce qu'ils n'auront pas reçu le soutien ponctuel nécessaire durant cette crise. Monsieur le ministre, quoi qu'il m'en coûte, je continuerai de me battre pour faire entendre leurs voix, en espérant que, un jour, ils auront la place qu'ils méritent.

Nous écoutons le ministre nous dire, comme il aime à le répéter pour développer son discours sur les finances publiques, que nous nous sommes endettés pour sauver notre économie et que cette « dette covid », nous devrons la rembourser. je souhaite le rappeler au Gouvernement, c'est lui qui a fait le choix politique d'un financement intégral par le déficit, donc par la dette. D'autres options étaient possibles, car l'on voit bien se dessiner le risque que l'on procède un dégonflement des dettes publiques par des politiques d'austérité réduisant les dépenses publiques et les politiques sociales. Cela se traduirait nécessairement par une chute de l'activité, donc une baisse des recettes fiscales ; par conséquent, le ratio de la dette par C'est au contraire par des ressources fiscales nouvelles qu'il faudrait aborder le sujet de la réduction de la dette, en privilégiant la taxation des hauts revenus, des hauts patrimoines et des entreprises multinationales, ainsi que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Doit-on évoquer l'actualité et le scandale des 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux obtenus par Apple, en Irlande, à cause du laxisme en matière de lutte contre les paradis fiscaux européens ?

rien ne justifie que ce type de revenu fasse l'objet d'un traitement avantageux. Ce sont autant de pistes que nous aurions aimé voir apparaître dans ce nouveau PLFR. Malheureusement, il n'en est rien. Nous aurons l'occasion d'en débattre au cours de l'examen du texte. Il faut Il faut relancer notre pays par le biais des territoires, de tous les territoires, c'est-à-dire par les territoires urbains, qui ont besoin de logements, de services, d'équipements et d'accompagnement dans la formation et l'emploi. Il s'agit donc de renforcer la politique de la ville.

Ils sont à même d'apporter les solutions aux problèmes que rencontre notre société, par leurs capacités d'accueil, les réseaux, les équipements et les services déjà présents et souvent souvent non saturés. Ils offrent également des réponses alternatives aux phénomènes de concentration, de saturation et de pollution qui touchent les territoires urbains. À cet égard, nous proposerons de voter le financement d'un nouveau programme, intitulé Villages du futur, pour favoriser le développement des villages constituant

ainsi indiscutablement à la cohésion des territoires. C'est aussi répondre aux attentes des populations urbaines souhaitant réaliser leur rêve de campagne, comme l'ont montré les flux de population lors du confinement. Il ne peut y avoir de relance de notre économie sans soutien, des dispositifs d'exonération fiscale et sociale, à nos zones rurales et aux entreprises qui souhaitent s'y installer et aux services qui y sont implantés. C'est le sens des amendements que nous défendrons, afin de proroger le bénéfice du classement en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les communes sortantes, jusqu'au 31 décembre 2021. Pour financer les actions à destination de ces territoires, pourquoi ne pas envisager des, afin d'orienter l'épargne locale en faveur de l'investissement dans les territoires ruraux ? mon intervention en évoquant deux sujets essentiels, insuffisamment pris en compte dans le projet de loi qui nous est soumis : la jeunesse et la transition écologique. transition écologique. Il y a urgence à répondre à la détresse des 700 000 jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi dans les prochaines semaines, ainsi qu'à l'angoisse de ceux qui basculent déjà dans la précarité. Le Président de la République a fait des annonces ce 14 juillet. Nous avons entendu

deux dispositifs, une « prime rebond premier emploi », pour toutes les entreprises qui embauchent un jeune, et une « aide rebond premier emploi », à destination des jeunes disposant de faibles ressources et en recherche d'emploi. En matière d'emploi, chaque jour, les plans sociaux tombent en cascade sur le pays, que ce soit au sein d'Air France, d'Airbus, d'Alstom ou de Sanofi ou d'entreprises plus modestes. Il devient urgent de réconcilier les différents acteurs de l'économie. Pour cela, nous avons besoin d'un nouvel esprit d'entreprise qui amplifie les efforts en faveur de plus de justice sociale, d'écologie et d'emploi. Il revient à l'État de n'accorder son soutien qu'aux entreprises qui poursuivent ces objectifs et qui renoncent à verser des dividendes à leurs actionnaires en 2020. Sur le plan de la transition écologique, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle doit être engagée rapidement, elle n'est toujours pas au programme du « monde d'après ». Dans les faits, est-il encore raisonnable de renflouer des multinationales polluantes, en toute opacité, sans contrôle démocratique, sans contraintes sans contraintes ni réelles contreparties exigées de leur part ? On ne peut injecter des dizaines de milliards d'euros dans l'économie et dans les entreprises, sous forme de prêts ou d'aides diverses, sans exiger des garanties pour le maintien de l'emploi et signer des engagements environnementaux Enfin, que dire du soutien à nos collectivités locales, qui sont les parents pauvres de ce budget, alors même qu'elles vont subir une perte évaluée à 7,5 milliards d'euros ? plus particulièrement les départements : après avoir assumé matériellement et financièrement les dispositifs de protection, on leur demande, dans l'urgence, de porter la responsabilité exclusive du financement des primes dont devrait légitimement bénéficier le personnel des Ehpad et des services à domicile. Les départements prennent également en charge l'accompagnement des personnes en difficulté. La réforme de l'assurance chômage fait peser sur eux un risque financier sérieux. De même, l'augmentation importante du nombre de nouveaux demandeurs d'emploi entraînera un accroissement du RSA qu'ils devront assumer.

Dans un récent rapport, le Haut Conseil des finances publiques recommande d'aider les collectivités à accompagner les acteurs locaux sur le terrain. Notre pays a besoin d'un investissement massif pour soutenir les communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux dans leurs projets de transition écologique sur divers thèmes- mobilités alternatives, rénovation énergétique des bâtiments publics, agriculture locale de qualité, économie circulaire notamment. Vous l'aurez compris, ce PLFR porte un plan de soutien inachevé du point de vue économique, social et écologique. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous espérons que les solutions que nous vous proposerons lors de nos débats retiendront toute votre attention et bénéficieront de votre soutien.

C'est le seul territoire français à continuer à être frappé de plein fouet et avec virulence par la pandémie. Les derniers chiffres, qui sont tombés aujourd'hui, sont très éloquents. Pour une Pour une population de 280 000 habitants, on compte 6 393 cas confirmés, avec un R0 oscillant entre 2,5 et 3,

Et le pic épidémique n'est prévu que pour la fin du mois ! Sur le plan économique, la situation est tout aussi inédite, avec un confinement qui n'a, en fait, jamais cessé depuis le 17 mars. En effet, le déconfinement de juin s'est vite traduit par un confinement ciblé, avec des restrictions sévères, comme la mise en quarantaine de quartiers et de villages ou Les conséquences sont dramatiques : nombreuses disparitions d'entreprises, augmentation du chômage, accentuation de la précarité, recul de l'activité de plus de 25 Aussi, si je salue les mesures déjà prises par le Gouvernement pour compenser les effets de la crise et celles qui sont proposées dans ce PLFR 3 pour les entreprises et les collectivités locales, la situation des collectivités de Guyane

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre des outre-mer ont pu s'en rendre compte lors de leur tout récent déplacement en Guyane. Élus locaux, syndicats, collectifs citoyens, socioprofessionnels, tous se sont mobilisés pour leur présenter des demandes légitimes et précises,

effet, nous avons la possibilité de redéployer un certain nombre de crédits. Surtout, nous disposons d'un projet de loi de finances rectificative de fin d'exercice, que nous utilisons traditionnellement pour adapter la fin de gestion. Cette dernière sera aussi l'occasion d'augmenter autant que nécessaire les crédits dont nous avons besoin. Nous veillons à ce que toutes les mesures qui ont été annoncées soient financées. Vous pardonnerez, j'en suis convaincu, mesdames, messieurs les sénateurs, le caractère non pas acrobatique, mais parfois un peu compliqué de ce financement. Nous nous adaptons à la crise, à ses conséquences et nous veillons à ce que les dispositifs qui ont été mis en place soient alimentés, pour qu'ils puissent être financés tout au long de la crise. Nous évoquerons également avec vous, pendant ce débat, le financement des mesures annoncées par le Premier ministre et le Président de la République, sachant que certaines d'entre elles feront l'objet de financements soit dans le cadre de la fin de gestion, soit au moyen de redéploiements. Je tiens à préciser, notamment pour rassurer celles et ceux qui s'inquiéteraient d'une impossibilité de financer les mesures de relance sur la fin de l'exercice 2020, que les premières mesures mises en oeuvre- je pense, par exemple, à la prime pour l'apprentissage -sont contenues dans ce PLFR et pourront donc être financées,

en considération le retard. Le PLFR de fin de gestion nous permettra de procéder à ces corrections. Nous ne le faisons pas à ce stade, considérant qu'il est trop tôt pour prendre de telles dispositions, mais nous travaillons toujours à la mise en oeuvre de la réforme des APL.

À aucun moment de l'histoire récente, les conséquences d'une crise n'ont été compensées auprès des collectivités sous forme de garantie de ressources. La dernière crise systémique que nous ayons connue, celle de 2008-2009, s'était traduite, pour les collectivités, par la possibilité

sera au minimum de 1 000 euros pour les collectivités bénéficiaires. Cependant, les collectivités dont les recettes, en 2020, seront égales ou supérieures à la moyenne de celles des trois années précédentes ne seront pas éligibles à un versement. Nous ne pouvons pas admettre la comparaison avec le fonds de solidarité et une forme de versement forfaitaire.

par rapport à l'adoption des dispositions par le Parlement. Ce n'est pas une formule totalement classique, j'en conviens bien volontiers, mais c'est la seule que nous ayons trouvée pour permettre aux collectivités de procéder aux délibérations,

que, lors de la dernière crise systémique de 2008-2009, les DMTO avaient diminué de 10 à 11 % la première année et de 25 % la deuxième année, mais qu'ils avaient augmenté de 30 % dès 2010 et de nouveau de 25 % en 2011. Autrement dit, l'inversion des cycles en matière de DMTO peut être extrêmement rapide, ce qui nous amène

Nous sommes effectivement dans une situation extrêmement particulière, avec une dette qui va atteindre 120 % du PIB et un déficit qui s'élève à 220 milliards d'euros,

qu'une partie sera mobilisée par Bpifrance et la Caisse des dépôts et qu'une partie pourra aussi être prise en charge dans le cadre du plan européen. Cela signifie que, si nous avions recours à la fiscalité pour financer ces mesures d'urgence et d'accompagnement, ce n'est pas un choc, mais un tsunami fiscal que subiraient les Français et les entreprises ! Si je suis

de la solidité et de la crédibilité de la signature de notre pays sur les marchés financiers. On peut nous reprocher d'être à leur merci, mais il faut aussi reconnaître que c'est sur les marchés financiers que nous trouvons les financements nécessaires pour pour répondre à la crise, mais aussi, plus généralement et plus traditionnellement, pour assurer le financement de l'État. Alors que nous empruntons encore aujourd'hui dans des conditions tout à fait favorables, l'une des lignes de conduite que nous devons observer consiste à garantir la crédibilité de cette signature, pour que les choses soient tenables. C'est ce qui nous amène, sur des crédits qui peuvent avoir un caractère récurrent, à nous en tenir à une certaine rigueur. C'est ce qui m'amène désormais, dans les relations que je peux avoir avec mes collègues pour la préparation du PLF pour 2021, à faire preuve de cette même attention à ce que la trajectoire pluriannuelle soit la mieux respectée possible. Monsieur

de lutte contre la crise, comme le fonds de solidarité, les prêts garantis, ou encore le dispositif plein et maximal de chômage partiel, soient prolongés, en Guyane, non pas jusqu'à une date butoir arrêtée par la loi, mais jusqu'au dernier jour du dernier mois au cours duquel nous aurons constaté l'état d'urgence, de manière que la durée de ces dispositifs soit

les indicateurs sociaux donnaient le signe qu'il faut agir. Je ne doute donc pas que je pourrai compter sur votre soutien sur un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment aux dispositions du projet de loi de finances rectificative qui tendent à soutenir soit l'embauche des plus jeunes, soit l'accompagnement des jeunes précaires, en particulier des étudiants. Je vous rejoins sur

La séance est reprise.

La République En Marche. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique. « D'ici à la fin de 2021, nous souhaitons que tous les territoires-

la ministre, acte 20 milliards d'euros pour la croissance écologique, dans l'optique de gagner la bataille pour le climat et la biodiversité, afin que l'économie française devienne la plus verte et la plus décarbonée d'Europe.

Madame la ministre, quelle sera la place des collectivités, en particulier des maires, dans ces politiques d'avenir ? Quel cahier des charges pour les contrats de développement écologique, avec quels financements ?

sont au coeur de notre vie quotidienne, plébiscitées par nos concitoyennes et nos concitoyens. La crise nous l'a rappelé très fortement. Nous devons y répondre.

et Social Européen. Ma question s'adresse à Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, et à M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports. Une politique de modernisation des infrastructures de transport au service de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement doit être intégrée au programme d'investissements publics de notre pays pour la prochaine décennie. Il faut rendre compatibles et complémentaires le développement économique, l'écologie et le désenclavement des territoires. La mutation des modes de transport en est un élément majeur. À côté du transport routier, auquel il manque quelques maillons, et du transport fluvial, dont le développement doit être accéléré- le canal Seine-Nord-Europe a pris beaucoup de retard -, se pose la problématique du transport ferroviaire qui constitue un levier essentiel de l'accessibilité des territoires et de la démarche écologique, cette dernière étant parfois- trop

contre 46 % en 1974, la moyenne européenne étant de 17 %. Cette faiblesse structurelle se caractérise par l'abandon de dessertes industrielles, aussi bien en termes d'approvisionnement que d'expéditions, et par l'affaiblissement de la capacité logistique de nos activités portuaires. En termes de fret ferroviaire, y compris pour le ferroutage, nous sommes à la traîne de l'Europe. Il s'agit pourtant d'un domaine créateur d'emplois et hautement stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à lancer sur dix ans un plan Marshall ferroviaire nécessitant plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements pour remettre notre pays à niveau et permettre de dégager une offre de service plus compétitive et plus écologique ?

voulu préserver les lignes aériennes d'aménagement du territoire selon une philosophie qui consiste à mieux articuler les modes de transport entre eux pour répondre aux spécificités des territoires et aux besoins de leurs habitants et de leurs entreprises, afin de garantir, comme vous l'avez souligné, leur attractivité. Nous allons encore accélérer. Le Président de la République et le Premier ministre ont eu l'occasion de s'exprimer récemment sur ces questions. Les transports seront au coeur du plan de relance. Nous poursuivrons la contractualisation avec l'ambition de sauver les 9 000 kilomètres de petites lignes ferroviaires. Nous voulons créer de nouvelles lignes de trains de nuit- vous avez mentionné cette ligne qui passe par Brive et Rodez. Nous avons pour ambition de doubler la part modale du fret ferroviaire, encore trop faible dans notre pays. Nous aurons l'occasion d'annoncer la création de nouvelles autoroutes ferroviaires prochainement.

pays. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, madame la ministre de la transition écologique, mes chers collègues, la Convention citoyenne pour le climat, créée sur l'initiative du président Macron, a formulé 149 propositions. Le chef de l'État avait promis la transcription de celles-ci dans la loi. Dès le 29 juin, il annonçait pourtant qu'au moins trois d'entre elles ne seraient pas retenues, dont la taxe de 4 % sur les dividendes. Et pourtant, point d'écologie sans solidarité ni justice sociale ! Le lendemain, Agnès Pannier-Runacher révélait que le moratoire demandé sur la 5G, luxe énergivore bien inutile dans un pays ne sont même pas desservis en totalité par internet, n'était pas non plus envisagé. Le 14 juillet dernier, le président Macron a certes parlé d'écologie- il est vrai que ce thème semble aujourd'hui pourvoyeur de voix. Annoncer des mesures déjà envisagées dès 2018, comme la rénovation thermique des écoles et des Ehpad, c'est faire du neuf avec du vieux. En revanche, combien de petites lignes ferroviaires sauvées ? Combien de tonnes de fret ferroviaire supplémentaires ? Il s'agit non pas d'opposer « croissance écologique » et « décroissance verte », mais de l'impérieuse nécessité de changer de modèle social et économique. À quand le référendum visant à inscrire dans la Constitution la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité ? À quand le projet de loi validant les propositions de la Convention ? Ferez-vous en 600 jours ce que vous n'avez pas fait en trois ans ? La

pour viol, harcèlement et abus de confiance concernant une sombre affaire d'échange de faveurs sexuelles contre une intervention à la Chancellerie. Ce que vous dites est scandaleux ! Depuis 2017, nous avons vu nombre de ministres démissionner suite d'affaires fiscales ou financières, ou encore pour consommation intempestive de homards ... Mais dans ce cas précis, rien : « circulez, il n'y a rien à voir ! » et rien à comprendre. Il n'y a pas de problème

Que nous dites-vous en réalité ? Que M. Darmanin est innocent, que la victime ment, au mépris des principes d'équité, du contradictoire et d'équilibre entre les parties. Pis, vous ignorez le conflit d'intérêts en puissance que représente cette nomination que se passera-t-il en cas de mise en examen d'un ministre qui sera l'autorité hiérarchique des policiers chargés d'enquêter sur ses agissements ? Que les députés LaREM se rassurent, il s'agit non pas de nier la présomption d'innocence, nous y sommes très attachés mais de vous interroger sur le signal délétère envoyé à toutes les victimes. Vous qui en appelez à l'exemplarité de la politique et à la lutte contre les violences faites aux femmes, quel message envoyez-vous aux Françaises et aux Français lorsque vous faites fi de la parole des victimes ? Mesurez-vous bien les conséquences de cette nomination ?

ce sont les principes fondamentaux de l'État de droit. Je suis ici en tant que chef du Gouvernement dans une assemblée parlementaire. M. Darmanin n'est pas mis en examen. M. Darmanin n'a fait l'objet d'aucune condamnation et, à ce que je sache, chaque fois que l'autorité judiciaire a eu à se prononcer dans cette affaire, elle a rendu des actes consacrant son innocence. M. Darmanin a droit au respect des principes de la République comme tous les citoyens.

du respect des principes fondamentaux de la République, que j'ai fait cette proposition. Votre intervention suppose donc

ou tués au cours de ces opérations. Nous avons payé un lourd tribut. Nous devons donc faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard de ce territoire. Le G5 Sahel est un soutien fondamental au coeur duquel se trouve le Mali,

du dialogue. Elle est bien évidemment aux côtés de ses ressortissants, à travers son ambassade, pour assurer leur sécurité, et aux côtés de ses partenaires internationaux pour appuyer une solution d'avenir.

l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle et la constitution d'un gouvernement de consensus. Le Premier ministre Cissé y travaille. Nous pouvons aussi noter avec satisfaction que celles et ceux qui avaient été arrêtés lors des débordements ont été libérés. Nous appelons le président Keïta à continuer dans cet esprit de responsabilité. Nous soutenons la nouvelle mission de la

Un sapeur-pompier, qui intervient sur un incendie de voiture, est la cible d'un tir par arme à feu et voit une balle lui traverser le mollet. Notre collègue Franck Marlin, maire d'Étampes, présent sur les lieux au moment de cette véritable tentative d'homicide, pourrait égrener les actes d'incivilité, de violence urbaine insupportable dont sa ville est victime depuis tant d'années, à l'instar de très nombreuses villes en France. Vous étiez hier sur place, à ses côtés, pour témoigner de votre soutien aux soldats du feu, ainsi qu'à l'ensemble des forces de l'ordre. Nous vous en remercions. Monsieur le ministre, je vous sais homme d'action et de responsabilité. Mais au-delà du dépôt de plainte systématique que vous avez appelé de vos voeux hier, ce qui constitue, reconnaissons-le, un strict minimum, comment comptez-vous sortir de la posture, des tweets et des discours creux auxquels votre prédécesseur nous a malheureusement trop souvent habitués durant cette triste première moitié de quinquennat ? Vous avez déclaré hier : « la République est partout chez elle ». Assurément, monsieur le ministre ! Dès lors, comment comptez-vous mettre hors d'état de nuire ceux qui n'ont pas cette idée de la France que nous avons en partage et qui est notre fierté nationale ? En d'autres termes, quand et comment comptez-vous sortir la France de la chienlit dans laquelle elle se trouve plongée ? C'est excessif ! La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

pour leur dire l'émotion qu'a suscitée non pas ce simple fait divers, mais cette attaque contre la République, contre les sapeurs-pompiers qui portent l'uniforme de la solidarité. L'un d'entre eux a été blessé par balle lors d'une intervention- somme toute banale -visant à éteindre un incendie de véhicule sur un parking.

Il va bien falloir que ce gouvernement fasse ce qui n'a jamais été fait en s'attaquant à ceux qui sont contre cette nation et qui n'ont plus rien à voir avec notre société républicaine.

lors des débats sur l'état d'urgence sanitaire, je vous interrogeai, ainsi que votre collègue Cédric O, sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à choisir Microsoft, l'un des Gafam, pour gérer les données de santé recueillies par la plateforme Health Data Hub, Cette décision a été prise à l'automne 2019 dans des conditions opaques, dénoncées par un collectif d'experts, sans appel d'offres, au détriment de toute entreprise française ou européenne. La réponse de Cédric O, arguant qu'il n'y avait aucune entreprise française capable de répondre aux exigences techniques de cette gestion, a été édifiante. Elle a d'ailleurs soulevé beaucoup de protestations dans les jours qui ont suivi. Depuis, les débats vont bon train. Je me réjouis qu'il y ait une prise de conscience,

peu protectrice. En l'état, monsieur le ministre, je vous poserai deux questions fondamentales, qui attendent des réponses politiques, et non techniques. Oui ou non les données des Français sont-elles un actif stratégique majeur, auquel cas elles ne sauraient être remises entre les mains d'acteurs étrangers ? Oui ou non allons-nous nous doter enfin d'une politique industrielle offensive permettant d'accompagner nos entreprises et appliquer la préférence communautaire, comme ont su le faire les Américains, créant l'écosystème que nous connaissons et dans lequel nous vivons aujourd'hui ?

investi, ces dernières années, quelques centaines de millions d'euros par an dans les technologies du numérique, là où les États-Unis investissaient plusieurs dizaines de milliards de dollars

il y a eu une phase de préfiguration au cours de laquelle il a fallu agir vite pour identifier un acteur capable de développer une plateforme de gestion et de sécurisation des données. Factuellement et juridiquement- le président de l'Anssi l'a d'ailleurs confirmé -, Microsoft est considéré, dans son entité gestionnaire des données de santé françaises, comme une entité européenne, même si le groupe est américain. Cela dit, oui, il y aura un appel d'offres : pour le fonctionnement pour le fonctionnement au quotidien et dans la durée de cette plateforme, nous serons amenés à faire appel d'offres. Il faut conclure. Et j'espère que nous pourrons identifier un grand acteur européen, voire, pourquoi pas, français, pour assurer dans la durée la gestion, le stockage et le partage de ces données. Ma question, monsieur le ministre, est on ne peut plus d'actualité, puisque nous apprenons aujourd'hui que, considérant que les risques d'ingérence des services de renseignement américains sur les données des Européens étaient trop importants, la Cour de justice de l'Union européenne vient d'invalider l'accord de transfert des données dit. Et Microsoft obéit bien à la législation

Après avoir assuré la continuité pédagogique, les professeurs ont donc été particulièrement attentifs à la demande de leur ministre de tutelle en se montrant bienveillants lors de l'examen des dossiers des candidats au baccalauréat. Certes on peut se réjouir de cette indulgence des jurys de délibération, mais le risque de dévaluation du diplôme n'est quand même pas très loin

accueillir davantage de monde dans des locaux exigus construits il y a plus de quarante ans ; appliquer des règles sanitaires de distanciation sociale pour éviter la propagation du virus ; proposer des modules de remédiation pour tenir compte d'une année scolaire qui a été très largement tronquée. Madame la ministre, que proposez-vous aux établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre de faire face à ces lourdes contraintes ?

L'immense majorité d'entre eux a eu néanmoins le courage de continuer à suivre des enseignements dans des conditions de confinement extrêmement difficiles à vivre pour l'ensemble de nos concitoyens, et plus particulièrement pour les jeunes. Permettez-moi aussi de saluer le travail de tous les enseignants qui les ont accompagnés. Oui, vous avez raison, cette année, l'ensemble de ces jeunes : ceux qui vont entrer dans l'enseignement supérieur, ceux qui désireront poursuivre leurs études, et ceux qui vont entrer sur le marché du travail. Et nous savons que ce sera compliqué. C'est pourquoi le Président de la République, le 14 juillet, et le Premier ministre, hier, lors de son discours de politique générale, ont indiqué que notre priorité serait de trouver une solution pour chacun de ces jeunes. Vous le savez, puisque vous avez tous, ici, participé à la construction de la loi Orientation et réussite des étudiants : nous avons des outils à cette fin. Plus d'un milliard d'euros sont investis dans le plan Étudiants, et des outils ont été créés par les établissements pour accompagner les jeunes et les prendre tels qu'ils sont de manière à les amener vers la réussite. Quant à la plateforme Parcoursup, elle a fait la preuve de sa robustesse

des lycéens ont reçu une proposition, et nous sommes en train d'en accompagner individuellement plus de 9 000. Nous avons travaillé à la création de plusieurs milliers de places en BTS, en filières courtes, en formations professionnalisantes, plus de 1 000 nouvelles formations en apprentissage, parce que nous devons aussi accompagner les jeunes qui ont besoin de l'apprentissage pour étudier. Nous trouverons une solution pour chacun de nos jeunes ; cet engagement a été pris au plus haut niveau. La parole Madame la ministre, je ne doute pas de votre volonté et de celle du Président de la République de régler ce problème. Néanmoins, nous avons un problème structurel. Les services du ministère

Le Gouvernement a d'ailleurs fait reposer en grande partie sa stratégie de gestion de la crise et de déconfinement sur les collectivités. Les élus locaux ont fait preuve de réactivité et d'adaptabilité, compensant certaines rigidités et imprécisions de l'État, et démontrant de nouveau l'importance des acteurs de proximité.

En plus de réduire leurs capacités de mobilisation, cette chute des ressources altère aussi leur agilité, alors que les collectivités seront amenées à jouer un rôle central dans le plan de développement économique annoncé. Je pense notamment à la relance de l'investissement et de la commande publique, pour cette année et pour 2021. Le troisième projet de loi de finances rectificative actuellement en discussion contient des mesures, à hauteur de 4,5 milliards d'euros, destinées aux collectivités- essentiellement des avances remboursables. Celles-ci viennent partiellement amortir le choc financier mais ces aides suffiront-elles à maintenir la capacité d'investissement des collectivités dans des secteurs décisifs tels que les mobilités, le déploiement du numérique, la relance verte ou la relocalisation d'activités stratégiques ? seront-elles en capacité de poursuivre leur action en faveur de l'égalité territoriale et de la justice sociale et de permettre aux territoires ruraux de relever le défi démographique par une politique d'accueil ? Plus globalement, n'est-il pas temps, madame la ministre, de libérer les collectivités de tout un ensemble de contraintes budgétaires qui réduisent leur autonomie fiscale et d'amorcer un virage ouvertement décentralisateur ? Pourriez-vous enfin nous préciser dans quelle mesure l'Agence nationale de la cohésion des territoires sera mobilisée pour accompagner tant les porteurs de grands programmes que les projets émergents locaux, dont le nombre devrait être multiplié en vue d'impulser la relance ?

plusieurs centaines de projets qui sont prêts à démarrer. Et, vous le savez, Territoires d'industrie est animé par les régions, par les intercommunalités et par les chefs d'entreprise.

immédiate et à long terme, pour les collectivités territoriales. J'ajoute que les CPER comprennent un volet territorial qui concerne tous les niveaux de collectivités : les communes, les intercommunalités, les départements.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique. Dans la valse des milliards, qui finit par donner le vertige, les nouveaux crédits consacrés à l'écologie sont passés en une semaine de 15 à 20 milliards d'euros. Important en valeur absolue, certes, cet engagement annoncé ne représente pourtant qu'à peine 4 % des plus de 500 milliards d'euros de crédits débloqués par le Gouvernement. Malgré ces sommes, nous avons du mal à comprendre tant la cohérence de votre politique environnementale et écologique que vous êtes la quatrième ministre chargée de l'écologie en à peine trois ans. Haut Conseil pour le climat, Convention citoyenne, conseil de défense écologique ... : autant de paravents pour mieux masquer vos incertitudes et tenir à distance les propositions du Parlement. À ce stade, madame la ministre,

pour la réplique. En termes simples, je vous dirai que le disque est rayé et que les Français n'ont plus confiance. Le Premier ministre l'a lui-même expressément Pour développer la filière hydrogène, vous alignez 100 millions d'euros, quand l'Allemagne met plus de 10 milliards d'euros sur la table. Vous prônez une économie décarbonée sans rendre d'arbitrages clairs en faveur des énergies renouvelables, et vous affaiblissez notre filière nucléaire, acteur majeur de décarbonation.

comme la crise actuelle nous le rappelle. Vite, donc, au-delà de la « vélorution » magique post-covid, abandonnez la verticalité de vos politiques et faites de l'environnement le socle d'un nouveau pacte de confiance, reposant sur trois piliers, écologique, économique et social.

Dans le discours de politique générale de M. le Premier ministre qui nous a été lu hier, on retrouve le mot « territoire » à vingt-cinq reprises. Dans les mêmes phrases, on parle de « confiance », on parle d'« intelligence », on parle de « proximité Vous imaginez combien ici, au Sénat, nous sommes sensibles à tout cela. Notre pays a pu compter sur les collectivités territoriales pour gérer et assumer les charges de la crise sanitaire. Il aura besoin, demain, de ces mêmes collectivités pour panser les plaies et relancer la machine économique. Les conseils départementaux, avec leur compétence sociale, ont été inventifs ; ils ont essayé d'apporter une aide adaptée aux besoins les plus criants. Ainsi en est-il en Haute-Savoie, où les élus ont voté un dispositif d'aide à 1 600 entrepreneurs qui ont été très sévèrement touchés par la crise. À l'instant où je vous parle, le virement de ces aides, bien que celles-ci aient été considérées comme conformes au droit au terme du contrôle de légalité du préfet, n'est toujours pas effectif. Cette situation est pénalisante et suscite la plus grande des inquiétudes parmi les élus. Madame la ministre, sans attendre que la différenciation devienne un principe organique ou constitutionnel, comment entendez-vous permettre aux collectivités d'être de vrais acteurs de l'après-crise ?

a adopté un règlement d'aide en faveur des travailleurs non salariés ne bénéficiant pas du chômage partiel. Sa délibération a été transmise au préfet, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques pour qu'ils puissent en examiner la légalité. Et, vous le savez, le contrôle de légalité est un service à rendre aux collectivités. Ce contrôle a été effectué en lien avec le président du conseil départemental, qui a eu l'occasion de fournir toutes les informations utiles. À l'issue de cette instruction, dont je rappelle qu'elle est parfaitement normale dans un État de droit, il apparaît que le règlement adopté par le département institue bien une aide de nature sociale destinée à des personnes physiques et conditionnée à des plafonds de ressources.

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, à l'occasion de la traditionnelle interview du 14 juillet, le Président de la République a affirmé, avec assurance : « Nous avons réussi à endiguer le virus et à retrouver presque presque une vie normale ». En tant que médecin ayant exercé pendant la crise et en tant que parlementaire informée des remontées du terrain, j'ai l'impression que nous ne vivons pas la même réalité. Depuis plusieurs semaines déjà, les indicateurs nous alertent : le virus est toujours là et, dans certains départements, il progresse de nouveau, et façon très inquiétante. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas sortis d'affaire, loin de là, et le chemin vers la vie presque normale risque d'être beaucoup plus long qu'annoncé au vu des mesures que vous prenez trop tardivement, ou que vous ne prenez pas.

Notre président de groupe, Bruno Retailleau, a demandé ce matin l'application immédiate de cette mesure, et vous avez finalement entendu raison, mais quelle perte de temps ! Par ailleurs, des dépistages systématiques et massifs doivent être organisés régulièrement, car c'est bien là le moyen le plus efficace pour briser les chaînes de contamination. Nous avons le sentiment que vous n'avez rien appris : nous sommes dans la même situation qu'au mois de février, avec un virus qui reprend sa progression. Monsieur le ministre, face à l'urgence, le Gouvernement doit entendre l'inquiétude des professionnels de santé et adopter une stratégie offensive ; cette épidémie ne sera éradiquée que par des mesures drastiques. Ma question est donc la suivante

Merci, madame la sénatrice, pour cette question qui, comme on le dit en médecine- vous et moi sommes médecins -, a été posée avec tact et mesure. Laissez-moi vous féliciter sincèrement d'avoir repris la blouse pendant la période épidémique. Je pense que les Français vous en savent gré. nous entendre, madame la sénatrice, sur plusieurs constats. S'agissant d'abord du port du masque, qui sera rendu obligatoire dans les milieux fermés, vous soulevez la question du 1 août. Vous le savez, nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité des Français.

Néanmoins, madame la sénatrice, vous avez été entendue avant même d'avoir posé votre question, puisque le Premier ministre s'est engagé ce matin à ce que l'obligation soit entérinée dès la semaine prochaine. Je peux même vous dire que, en l'état actuel de la réflexion, nous nous dirigeons vraisemblablement vers une obligation à compter de lundi ou mardi, en tout cas du tout début

vous faire constater qu'un certain nombre de pays ont été conduits à un reconfinement territorial parfois généralisé, y compris des pays dont j'ai souvent entendu parler dans cet hémicycle, pendant la période épidémique, comme étant des modèles. Si cela n'a pas été le cas en France, c'est pour une simple raison, madame la sénatrice : pendant douze semaines, pendant douze semaines, les indicateurs se sont améliorés continuellement. En revanche, vous avez raison de souligner que certains indicateurs doivent nous alerter et nous inquiéter- je l'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale -, dans certains hôpitaux parisiens ou en Mayenne, notamment. C'est pourquoi nous démultiplions les capacités de tests et de. des heures durant pour expliquer pourquoi il était fondamental de ne pas désarmer juridiquement l'exécutif, le Gouvernement, dans sa capacité à agir et à prendre les bonnes décisions au bon moment alors que nous sortions de l'état d'urgence sanitaire. Je vous propose, madame la sénatrice, de relire les comptes rendus des débats : vous y verrez que je n'étais

Oui, mettre en place de telles mesures nécessite du temps ; mais vous auriez dû les prendre avant, et ne pas vous y résoudre au dernier moment. Soyez vigilant, monsieur le ministre : demain, lorsque la population sacrifiée et les familles vous demanderont des comptes, vous ne pourrez plus dire : « nous ne savions pas ».

par le Président de la République comme par le Premier ministre : la jeunesse est la priorité des mois qui viennent, car il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire la difficulté des jeunes à accéder à l'emploi.

Cette épreuve exceptionnelle appelle des décisions exceptionnelles, en particulier pour les quelque 700 000 jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Notre jeunesse, dans sa diversité, a plus que jamais besoin de perspectives d'avenir. Le meilleur des plans de relance, c'est celui qui ne laisse aucun jeune en plan C'est pourquoi des mesures ambitieuses sont très attendues. Nous examinerons demain le troisième budget d'urgence, dans lequel figurent, notamment, une prime à l'embauche exceptionnelle pour le recrutement des apprentis, allant jusqu'à 8 000 euros, ou bien une prime de 200 euros pour les jeunes les plus précaires.

la bonne application de ces mesures dans les territoires sera la garantie du succès de cette démarche. Dès lors, madame la ministre, et sans préjuger ce que sera la concertation avec les partenaires sociaux, quels sont les objectifs, les axes, le calendrier

Pour les jeunes souhaitant s'engager sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, nous devons veiller à ce qu'ils puissent trouver une entreprise d'accueil. C'est ce que nous faisons en prévoyant une prime de 5 000 euros pour les moins de 18 ans, 8 000 euros pour les autres. Nous allons donc continuer à mettre le paquet sur l'apprentissage. nous créerons 100 000 services civiques supplémentaires, pour permettre à des jeunes de s'engager dans des missions utiles à la société en attendant une conjoncture meilleure. Pour les jeunes les plus en difficulté, 300 000 parcours ou contrats d'insertion supplémentaires

nous préparons, avec les partenaires sociaux, avec les territoires, avec les parlementaires, une réponse à la hauteur des enjeux et de l'alimentation. Au mois d'août 2016, le Gouvernement oeuvrait pour l'interdiction, à compter du 1 septembre 2018, de certains produits sanitaires, fongicides et insecticides, dont, d'ailleurs, la non-dangerosité sur l'homme a été prouvée.

Que fait le Gouvernement ? Il est en train de ruiner les cultures françaises, en particulier celle de la betterave, qui se trouve atteinte par une invasion de pucerons lui transmettant la jaunisse virale, avec des pertes colossales à la

Si les bonnes dispositions ne sont pas prises d'ici à quinze jours, il n'y aura plus d'alcool- plus de gel hydroalcoolique -, plus de sucre, plus d'alimentation pour le bétail ! Les Français consommeront alors des produits importés et fabriqués avec les substances Est-ce ainsi que l'on dynamise une filière qui fonctionne ? Voulez-vous l'anéantir ? Quelle est votre solution ?

Le temps nous presse, monsieur le ministre. Le Président de la République, lors de son allocution, a de nouveau affirmé qu'il fallait réapprendre à produire ce dont on a besoin. Vous-même, monsieur le Premier ministre, vous affirmiez hier que nous sommes trop dépendants de nos partenaires extérieurs. Je prends acte de vos propos et, en même temps, de vos contradictions. Aussi, je le dis avec force, j'accuse le Gouvernement de la destruction de la filière betterave. J'accuse le Gouvernement de la destruction de la filière alcool et de la fragilisation de notre production d'énergie et d'aliments pour le bétail. Une attitude semblable est incompréhensible pour notre société et pour le monde agricole, déjà au bord du gouffre. Faites vite, monsieur le Premier ministre

Dans le contexte présent- suppression des deux tiers de lits en psychiatrie, insuffisance des accueils alternatifs et des équipes mobiles, financement sans lien avec les besoins locaux, accès difficile aux centres médico-psychologiques, 20 % des postes du secteur public non pourvus,

Pendant le confinement, les pertes de suivi, les ruptures de traitement ont concerné 10 % des malades. Faute de moyens humains suffisants, ont été mises en oeuvre des privations de liberté injustifiées sur le plan médical et illégales, dans des conditions indignes pour les malades. de privation de liberté, attire l'attention sur la question des droits des patients, sur l'enfermement de plus en plus important des malades mentaux. Elle s'interroge sur les nouvelles règles des hospitalisations sans consentement, sur l'utilisation abusive de l'isolement et de la contention.

avec les Français. Pendant toute la période de crise épidémique, des soutiens psychologiques ont été mis en place par des associations et des professionnels du secteur sanitaire et médico-social, y compris, d'ailleurs, à destination des soignants eux-mêmes, qui ont été soumis à un stress

monsieur le ministre, qui me touchent particulièrement. L'engagement et le dévouement des soignants ne sont pas mis en doute,